Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici de nouveau réunis pour discuter devant votre assemblée du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental Sur les quinze articles de ce texte, sept ont été définitivement adoptés. En effet, plusieurs modifications d'importance proposées par le Sénat ont été entérinées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement, notamment en matière de déontologie. Après des débats si complets en première lecture, il n'est plus nécessaire, je le crois, d'exposer de nouveau le détail de ce projet de loi organique qui a pour ambition de réformer le CESE, réforme que nous nous accordons tous à considérer comme nécessaire. Je parle d'ambition, car ce ce projet de loi organique propose effectivement une réforme ambitieuse pour le CESE. Je pense par exemple à la possibilité qui sera offerte à de jeunes citoyens en devenir de prendre part à la réflexion et au débat publics, avec l'ouverture du droit de pétition à partir de l'âge de 16 ans. Mais je voudrais aujourd'hui revenir plus précisément sur les points qui restent en débat et qui ont conduit votre commission à déposer une motion tendant à opposer la question préalable. En premier lieu, ce projet de loi organique, en prévoyant la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort, ne menace en rien la démocratie représentative. Je l'ai déjà dit, il n'y a ni confusion ni encore moins concurrence entre, d'une part, l'intérêt de recueillir l'avis de citoyens tirés au sort et, d'autre part, l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation élus au suffrage universel et qui, seuls, ont la légitimité démocratique. Renforcer la démocratie participative, ce n'est pas affaiblir la démocratie. Je crois au contraire que, plus nos concitoyens seront associés au débat public, plus la légitimité de ceux qu'ils éliront sera renforcée. C'est le voeu des Français, exprimé à maintes reprises ces dernières années. Nous devons les entendre. Par ailleurs, et la commission l'a elle-même mentionné, le CESE a déjà eu l'occasion par le passé de procéder à des consultations, en recourant au tirage au sort. Pour autant, et que je sache, cela n'a pas suscité chez nos concitoyens de remise en cause de l'exercice du droit de vote pour élire leurs représentants. En second lieu, l'article 6 du projet de loi organique, qui donne un effet substitutif à la consultation du CESE, ne va affaiblir en rien les études d'impact. Nous sommes tous d'accord pour dire que le CESE n'est pas assez consulté, que ce soit par le Gouvernement ou d'ailleurs par le Parlement. Il nous semble que l'une des raisons qui expliquent ce délaissement est la multitude d'organismes consultatifs, qui sont autant de concurrents pour le CESE. En accordant une place prépondérante au CESE, en cohérence avec celle qu'il tient dans nos institutions républicaines, nous allons lui redonner de l'attractivité. Et cela ne va en rien nuire à la richesse des consultations ou à la clarté de la répartition des compétences entre les différents organismes consultatifs. Tout d'abord, nous avons la chance, avec le CESE, de regrouper, au sein d'une même institution, des profils et des compétences extrêmement variés qui seront pleinement de nature à assurer un avis d'une grande richesse, comme c'est d'ailleurs déjà le cas. Ensuite, les discussions que nous avons eues en première lecture ont permis d'affiner le périmètre de l'effet substitutif de la consultation du CESE, tout en préservant la consultation d'instances éminentes comme le Comité des finances locales. la commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté en nouvelle lecture une autre garantie qui me paraît essentielle : le CESE pourra toujours consulter, dans le cadre de l'élaboration de ses avis, les instances consultatives compétentes. L'expertise de ces divers organismes pourra donc nourrir les avis du CESE et enrichir nos réflexions sur les projets de loi concernés. Pour toutes ces raisons, je crois que cette nouvelle rédaction de l'article 6 est de nature à atteindre nos objectifs, tout en répondant à vos craintes. L'autre grand sujet de discussion que nous rencontrons concerne la composition du CESE. D'abord, je m'inscris en faux avec l'analyse qui consiste à dire qu'en diminuant le nombre de membres du CESE, on l'affaiblirait.

avis d'un comité consultatif. Ces modifications permettent d'atteindre un équilibre entre tous les intérêts représentés. La représentation de nos outre-mer au sein du CESE suscite par ailleurs, je le sais, une attention toute particulière et bien légitime de la part de votre assemblée. Je voudrais ici essayer de vous rassurer quant aux garanties qui ont été apportées. Si le CESE ne représente pas les outre-mer, en revanche, la représentativité équilibrée de l'ensemble des composantes économiques et sociales de notre pays implique que les outre-mer y soient suffisamment représentés.

dans la troisième catégorie de membres du CESE relative notamment à la cohésion territoriale et en proposant une représentation des outre-mer à huit membres compte tenu des différents équilibres en cause. Cette nouvelle rédaction nous semble parvenir à un compromis équilibré. Si j'ai bien conscience que nous n'aurons vraisemblablement pas l'opportunité de discuter de nouveau du fond de cette réforme, voilà les points que je tenais à souligner devant vous aujourd'hui. Et si vous me permettez de regretter l'absence d'accord sur la réforme d'une institution constitutionnelle, permettez-moi également,

la baisse du nombre de membres du CESE. Pourquoi 25 % ? La réponse qui nous a été apportée est que le Président de la République en a décidé ainsi ...

La démocratie, c'est soit la population qui s'exprime directement, soit la population qui choisit des représentants. Une fois élus, ces derniers

M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notre démocratie vit une crise de confiance majeure.

Nous restons déçus du péché originel de ce texte : à droit constitutionnel constant, les possibilités pour le CESE de prendre toute sa place seront forcément limitées. Seule une réforme constitutionnelle nous aurait permis d'atteindre un niveau adéquat de transformation, pouvant inscrire dans le marbre pour le long terme le renforcement de la participation des citoyens et de la société civile. Jusqu'à présent, le CESE est très peu visible, trop peu écouté et rarement pris en compte dans la fabrique de la loi. Pourtant, la tenue de la Convention citoyenne pour le climat a montré l'engouement que pouvaient susciter chez les citoyens les démarches de démocratie participative.

Le maintien de la procédure simplifiée reste une erreur et ne va pas dans le sens du long terme ni d'une réflexion approfondie que nous souhaitons pour le CESE. Nous proposions la suppression complète de cette disposition, très peu utilisée et sans réelle efficacité. Ce texte contient donc des reculs, mais il est également porteur d'innovations bienvenues. Je veux ici parler du tirage au sort qui, pour nous, est un moyen utile de compléter la démocratie représentative et de revitaliser le débat démocratique. Cette procédure ne nous paraît pas, contrairement à ce qui a pu être avancé dans cette assemblée et en commission, mener à une « démocratie de la courte paille ». Nous appuyer, pour mener à bien notre mission de législateur, sur des assemblées de citoyens tirés au sort représentant une diversité de points de vue vient, selon nous, enrichir le processus de concertation et de prise de décision et renforcer notre légitimité de parlementaire par la création d'une confiance renouvelée avec les citoyens.

Nous saluons donc le processus de consultation par tirage au sort et de participation de personnes tirées au sort aux commissions du CESE. Nous soutenons également les dispositions visant à faciliter la saisine du CESE par voie de pétition dès l'âge de 16 ans, et ce sans critères géographiques. Enfin, nous souhaitons par ce texte renforcer la place des enjeux environnementaux au sein du CESE. Vous le savez toutes et tous, mes chers collègues, ces enjeux sont de plus en plus présents dans nos vies. Les effets du changement climatique se font très concrètement ressentir aujourd'hui : tensions sur l'utilisation de la ressource en eau, difficultés agricoles, augmentation du nombre et de accélération de la perte de biodiversité, etc. Dans ce contexte d'urgence climatique et écologique, renforcer la place des acteurs de la protection de la nature au CESE nous semble relever du simple bon sens.

Nous ne le déplorons pas sur le fond, puisque ce texte intègre certains apports utiles du Sénat, ainsi que des dispositions qui nous apparaissent toujours très bienvenues pour redonner au CESE la place qui lui revient aux termes de la Constitution. Ces dispositions sont aussi de nature à faire du CESE le « carrefour des consultations publiques » et de la participation citoyenne. Nous pouvons toutefois le regretter sur la forme. Je ne m'attarderai pas sur le constat, partagé sur toutes les travées, du déficit de visibilité de cette assemblée consultative, qui ne fait pas justice à la qualité de ses travaux. La proportion croissante des autosaisines- elle atteint 80 % en 2020 -parle d'elle-même. À ce titre, plusieurs dispositions ont fait l'objet d'un accord à l'issue de la première lecture entre les deux assemblées. Elles manifestent un objectif partagé d'accroissement du nombre de saisines du CESE et de renforcement de sa capacité à y répondre. Je pense à l'article 5 relatif à l'extension de la procédure simplifiée pour l'adoption des avis. Je pense également aux articles relatifs à la déontologie des membres du CESE, dont notre rapporteure a parfait la rédaction en première lecture. S'agissant du renforcement de la saisine du CESE par voie de pétition, les deux chambres ont consenti non seulement au dépôt des pétitions par voie électronique, mais également à la faculté, pour les mineurs de plus de 16 ans, d'en être signataires. monsieur le garde des sceaux, à cette disposition, animée par l'ambition de préparer ce groupe d'âge à l'exercice de sa citoyenneté. D'autres dispositions sont marquées par un désaccord de fond ; je pense aux articles 4, 6, 7 et 9.

À la différence du projet de loi organique initial, la rédaction actuelle maintient une garantie chiffrée sur la représentation des outre-mer au titre de la cohésion sociale et territoriale, présente dans le droit en vigueur et que notre Haute Assemblée avait utilement rétablie. Je salue cette garantie spécifique, dérogeant au renvoi à un décret opéré pour la composition des autres catégories. Bien sûr, nous pourrions discuter du chiffre, ramené à l'Assemblée nationale de onze à Il est proportionnel à la réduction globale de 25 % du nombre de membres. Et vous l'aviez rappelé, monsieur le garde des sceaux, il reste sans préjudice de la présence de représentants des outre-mer au sein d'autres catégories. J'y serai bien sûr attentif et le comité de suivi rétabli à l'Assemblée nationale n'apparaît, en ce sens, pas dénué d'intérêt. Pour terminer, je ne peux qu'exprimer un regret sur le désaccord de principe, acté par notre rapporteure dès le commencement des débats, sur la question du tirage au sort. Il a été dit que l'inscription dans la loi organique de ce procédé fragiliserait les fondements de notre démocratie et, pire, qu'il acterait l'avènement d'une « démocratie de la courte paille ». Pourtant, il n'est en aucun cas question de substituer des membres tirés au sort aux représentants de la société civile. Il ne s'agit pas non plus, puisque le caractère consultatif est bien précisé, de substituer le tirage au sort à la légitimité de l'élection qui, seule, peut asseoir par le mandat la décision souveraine. Nous regrettons ce point de crispation initial, qui a d'ailleurs animé nos débats. S'agissant des consultations publiques, une position commune aurait pu émerger. Il nous apparaît que, plus que le seul procédé, c'est la question du processus qu'il faut examiner. Les garanties procédurales, renforcées à l'Assemblée nationale par la nomination de garants, conforteront la pertinence et la qualité de cette participation citoyenne. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI s'opposera à la motion déposée par la rapporteure.

Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, annoncée dès juillet 2017 comme l'un des chantiers institutionnels majeurs du Président de la République, la réforme du Conseil économique, social et environnemental devait laisser place à la « Chambre du futur à un « trait d'union entre le monde politique et la société civile ». L'attente suscitée par le Gouvernement laissait penser que nous aurions à débattre de propositions novatrices, que la réforme de 2008 serait à reléguer au rang de simple dépoussiérage avant la grande rénovation de 2020.

Face aux critiques récurrentes qui lui sont adressées, je m'accorde avec vous, monsieur le ministre, sur la nécessité de la réformer pour que son travail puisse être nourri par une plus grande participation citoyenne, et ainsi reconnu à sa juste valeur. Mais pensez-vous pouvoir construire une « chambre pour et par la société civile », pour reprendre vos propos, en vous attachant à multiplier le nombre de pétitions et à systématiser la pratique du tirage au sort ? Le pouvoir démocratique d'une pétition ne réside pas dans le simple fait d'interpeller directement une institution décisionnelle et d'avoir, rapidement, une prise de position de cette dernière. C'est le débat que la pétition réussira à imposer sur le devant de la scène publique qui fera d'elle le garant efficace de la décision démocratique. Pour cela, elle doit coller à notre réalité nationale, et les critères de représentativité géographique et temporelle proposés par la commission des lois auraient permis de s'en assurer.

Dans un système représentatif comme celui de la France, nous devons tenter de renforcer la participation citoyenne en encourageant des actions responsables, dont nos compatriotes pourraient avoir l'initiative, et non en demandant leur avis à des citoyens qui n'ont pas été désignés par leurs pairs pour prendre la parole en leur nom. Nous soutenons néanmoins la simplification de la subrogation de la consultation des avis exprimés dans le cadre de l'élaboration d'une loi. Le CESE a la capacité de recueillir ces avis émanant d'instances représentatives locales et d'en faire la synthèse. De plus, le RDSE se réjouit de la suppression conforme de l'article 2. Comme nous l'avons exprimé lors de la précédente lecture, nous estimons que le contrôle de l'application des lois fait partie des prérogatives du Parlement depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Permettre à une minorité de parlementaires de requérir l'aide du CESE en demandant un avis sur la bonne application de la législation ne nous semble pas utile, mais plutôt redondant. Quant à l'organisation du CESE, nous soutenons le remplacement des personnalités qualifiées du collège 4 par des personnalités extérieures directement nommées par le Gouvernement. Elles pourraient être mobilisées au coup par coup sur un sujet particulier, pour plus de pertinence, et donc d'efficience. Au nom de mon collègue Stéphane Artano, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, je tenais aussi à vous faire part de nos inquiétudes quant à la représentativité de nos territoires d'outre-mer au sein du CESE. J'espère que vous aurez à coeur, monsieur le ministre, de corriger cet écueil. Enfin, je déplore que les relations des entités régionales que sont les Ceser avec le CESE restent inchangées et qu'il n'y ait eu aucune recherche de synergie. La prise en compte des territoires et de leur représentation est décidément bien difficile pour les gouvernements successifs du Président de la République ... Les membres du groupe RDSE sont en total accord avec le travail mené par la commission des lois du Sénat pour tenter d'enrichir ce texte.

comme on a pu l'observer à travers d'autres décisions concernant le paritarisme. Pour nous, c'est une fragilité démocratique. En revanche, à la différence de nos collègues

je voudrais revenir sur deux points de vigilance à l'égard du texte qui sera adopté et insister sur une interrogation véritablement légitime.

l'institution incarne une démocratie plus participative, plus moderne, plus mature, plus efficace. Tout est dit, il n'y a plus qu'à faire ! Le Sénat, en première lecture, a fortement enrichi le texte, 21 amendements ayant

la saisine des conseils consultatifs créés auprès des collectivités locales ou des groupements par le CESE à l'obtention préalable d'un accord des collectivités et des groupements concernés.

Le Sénat a souhaité également que les pétitions ne portent pas exclusivement sur des sujets locaux. Il a ajouté un critère géographique et porté de six mois à un an le délai pour se prononcer sur celles-ci.

Second point de vigilance : l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qui permet au Gouvernement, lorsqu'il consulte le CESE sur un projet de loi, de s'exonérer des autres consultations préalables.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un pays qui débat souvent de façon conflictuelle d'un certain nombre de sujets,

qui accompagne nos réflexions, que ce soit sur les conditionnalités indispensables en matière climatique et environnementale dans le plan de relance, sur la manière de vivre avec la dette, sur l'évolution d'une fiscalité qui pèse de plus en plus sur les revenus faibles et moyens, sur la place de la jeunesse dans la société, sur l'accélération de la révolution numérique engendrée par la pandémie, ou encore, alors que le projet de loi sur le séparatisme est lancé, sur le financement des cultes, l'évolution des obligations scolaires ou la liberté d'association. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, nous avons un gros désaccord avec la majorité sénatoriale sur l'article 4. Comme M. Benarroche l'a dit, nous croyons qu'il faut réformer, expérimenter de nouvelles choses, parce que la démocratie représentative est en crise. La démocratie représentative « à la grand-papa », c'est fini ! La révolution numérique a balayé le fonctionnement des partis politiques tel que nous le connaissions depuis des années. Les démocraties vont mal. Nous avons besoin de trouver de nouvelles manières de faire participer les citoyens à la décision, tout en restant très attachés à ce que ce soit l'élection qui confère la responsabilité de décider.

par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture sur la base d'un constat que nous partageons tous : il est nécessaire de réformer cette institution, qui, depuis longtemps, peine à trouver sa place dans notre système institutionnel. Cette assemblée, depuis plusieurs années, ne remplit plus véritablement la mission qui lui a été confiée par le constituant, à savoir représenter un trait d'union entre la société civile organisée et les pouvoirs publics, à tel point que nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'utilité du CESE ou qui plaident en faveur de sa suppression. Concurrencé par d'autres instances consultatives, qui disposent d'une capacité d'expertise plus spécifique sur des sujets d'une grande complexité, le CESE s'autosaisit de la plupart de ses sujets d'étude, faute de consultations externes, ce qui peut poser question pour une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 30 octobre dernier, a toutefois échoué à proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Parmi les points sur lesquels nos deux assemblées convergent, et qui se retrouvent dans le texte que nous examinons aujourd'hui, je citerai le maintien de la suppression des personnalités qualifiées dans la composition du CESE, proposé à l'article 7, ce qui conférera au collège des membres une plus grande légitimité. Néanmoins, nous divergeons sur des sujets essentiels. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité conserver la légitimation du tirage au sort dans le fonctionnement du CESE, actant ainsi un désaccord profond avec le Sénat. L'Assemblée nationale a également maintenu sa position en fixant l'effectif du CESE à 175 membres. Je déplore cette réduction de 25 % des effectifs du Conseil, qui n'apparaît reposer sur aucun critère objectif. De surcroît, cette diminution semble paradoxale, alors que la réforme vise à les solliciter davantage. ont précisé que les outre-mer ne disposeraient que de huit sièges, alors que le Sénat souhaitait leur en attribuer onze, afin que chaque territoire ultramarin puisse être représenté au sein du CESE. Concernant la question des règles déontologiques, le CESE ne peut demeurer la seule institution dont les membres sont exemptés des obligations déontologiques en matière de prévention des conflits d'intérêts. Aussi, je me réjouis qu'en nouvelle lecture l'Assemblée nationale ait repris l'essentiel des propositions du Sénat, concernant, notamment, la définition des conflits d'intérêts, les prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ou encore les souplesses laissées au CESE dans l'organisation de son dispositif déontologique. La seule divergence concerne concerne la réintroduction par les députés du rapport annuel d'activité des membres du CESE, dont nous pouvons douter de l'utilité. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si le CESE est une institution ancienne, paradoxalement, il demeure aujourd'hui une instance consultative méconnue, qui a encore du mal à exister. Il fait l'objet de critiques récurrentes en revenant, de temps en temps, sur le devant de la scène, dans le débat public ; ses travaux manquent de visibilité. Loin d'en faire une « Chambre du futur », ce texte demeure malheureusement en deçà des attentes que les annonces du Président de la République avaient. Beaucoup trop d'éléments entraînent de fortes réserves de notre part. Aussi, le groupe Les Indépendants s'abstiendra sur ce texte.

nous entamons cette semaine par le nouvel examen du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Cette nouvelle discussion a malheureusement été rendue nécessaire par l'échec de la commission mixte paritaire du 30 octobre dernier. Disons-le d'entrée de jeu, notre groupe ne rejette aucunement l'idée de rénover le CESE. Cet organe constitutionnel consultatif a un rôle à jouer afin de favoriser le dialogue entre les forces vives de la Nation et d'appuyer le législateur dans son travail. D'ailleurs, lors de la première lecture, notre rapporteur, Muriel Jourda, avait mis en exergue la sous-utilisation du potentiel du Conseil, tout en rappelant que, évidemment, il n'avait pas vocation à devenir une « troisième chambre ». De toute façon, le choix fait par le Gouvernement de réformer le CESE à droit constitutionnel constant écarte d'emblée toute possibilité de changements radicaux. Quoi qu'il en soit, il est devenu manifeste, au cours de la navette, que la vision du Sénat quant à l'avenir du CESE n'était pas entièrement partagée par la majorité et le Gouvernement. Cela dit, il convient de saluer, comme l'a fait le rapporteur, la qualité du dialogue qui a été noué dans le cadre de la recherche d'un compromis, dialogue qui a rendu possibles certaines convergences sur plusieurs sujets du texte. C'est ainsi que nous pouvons nous féliciter de voir que les députés ont maintenu les apports sénatoriaux relatifs à l'organisation interne du CESE. Il en va de même pour la structuration d'un dispositif déontologique solide, qui fera intervenir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, ces convergences ne peuvent masquer les points de désaccord substantiels qui persistent sur un certain nombre des principales dispositions du texte. Il en est ainsi de la question du recours au tirage au sort pour la participation des groupes de citoyens aux travaux du CESE. L'introduction d'un tel processus dans le fonctionnement d'une institution constitutionnelle, même consultative et dans le cadre d'une procédure de portée limitée, nous semble incompatible avec notre modèle de démocratie représentative. Quand bien même cela ne suffirait pas à nous dissuader, il ne faut pas oublier que, le jeu des récusations aidant, constituer un échantillon un tant soit peu représentatif par le biais du tirage au sort est quelque chose de passablement difficile, comme a pu le rappeler Philippe Bas à l'occasion de la CMP. Un autre point de désaccord majeur se situait au niveau du dispositif dit de « subrogation », à l'article 6 du projet de loi organique. Ce dernier permet au Gouvernement d'être dispensé de certaines consultations d'organismes, pourvu qu'il consulte le CESE. Si nous partageons évidemment le désir de donner corps au rôle consultatif du Conseil, il est simplement incohérent et inefficace de le faire de la sorte : d'une part, le CESE ne dispose pas des moyens techniques et administratifs appropriés d'autre part, une telle mesure risquerait d'abîmer simultanément sa légitimité, par défaut d'expertise technique, et celle des organes subrogés, qui se verraient ainsi dépossédés périodiquement de leur rôle. il y a d'autres dispositions problématiques sur lesquelles un accord n'a pas été possible. C'est le cas de la consultation des Ceser par le CESE et de la réduction des effectifs du Conseil, laquelle intervient au détriment des conseillers ultramarins.

défavorable à cette motion. Mais comme j'ai cru comprendre que je n'avais pas l'ombre de l'once d'une chance de vous convaincre de quoi que ce soit, et comme je n'ai, par ailleurs, pas le goût de l'effort inutile, je me rassois immédiatement.

Le scrutin est ouvert.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur,

j'ai eu l'occasion de le voir lors de l'examen de la mission « Sécurités » du projet de loi de finances pour 2021, le Parlement est très attentif aux dispositions qui permettent de mieux protéger les Françaises et les Français. Trois ans après l'adoption de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite « loi SILT », les dispositions qui ont été adoptées pour sortir de l'état d'urgence restent pleinement d'actualité. Il s'agissait de maintenir un niveau extrêmement exigeant de sécurité pour les Français, car la menace reste prégnante et la lutte contre le terrorisme demeure une priorité de l'action du Gouvernement. Pour cela, la loi SILT a mis en place des outils nouveaux, mais adaptés, garantissant un équilibre entre efficacité de l'action antiterroriste et préservation des libertés. Nous avons collectivement conscience du niveau extrêmement élevé de la menace qui continue à peser sur notre pays. L'attaque terroriste devant les anciens locaux de, celle de Conflans-Sainte-Honorine et celle de Nice montrent, si cela était nécessaire, que nos efforts ne doivent pas se relâcher et que nous devons continuer d'agir avec la plus grande détermination contre le terrorisme islamiste. Depuis 2017, quatorze attaques ont abouti sur le territoire national. Mais il faut aussi dire que, depuis 2017,

La loi SILT a permis à ces services de continuer à disposer, après la fin de l'état d'urgence, d'un cadre législatif efficace et adapté à leur action. Je souhaite cependant insister sur l'usage qui a été fait de ces outils nouveaux. Au 11 décembre 2020, 605 périmètres de protection ont été mis en place et huit lieux de culte ont été fermés. Dans le même temps, 370 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été notifiées- parmi elles, 63 sont actives à ce jour -et 397 visites domiciliaires ont été réalisées.

mesures. Il a également été rendu destinataire, chaque année, d'un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi. De la même manière, le Gouvernement a fait un usage raisonné de la technique dite « de l'algorithme ». Ainsi, depuis 2015, trois traitements automatisés ont été autorisés par le Premier ministre, après avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement La délégation parlementaire au renseignement a été rendue destinataire d'un rapport classifié au niveau « confidentiel défense », qui décrit la nature de l'apport opérationnel de ces traitements automatisés. Les mesures dont il vous est proposé de prolonger l'application par le présent projet de loi constituent donc des outils opérationnels indispensables pour les services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Il est important de outils ont été mis en oeuvre sous le contrôle attentif du juge, judiciaire et administratif, et, pour certains d'entre eux, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, avis que le Gouvernement a toujours suivis. Ils font l'objet d'un échange permanent avec le Parlement, sous la forme d'une information en temps réel et d'une évaluation régulière, que le Gouvernement a strictement respectées. Ces dispositifs ont démontré toute leur pertinence dans la prévention de la menace terroriste.

pérenniser dès à présent ces dispositions serait passer l'occasion de les adapter pour qu'elles répondent au mieux aux besoins des services, tout en respectant l'équilibre qui a présidé à leur adoption. Le Gouvernement envisageait par ailleurs, avant l'émergence de la crise sanitaire, de soumettre au Parlement avant l'été un projet de loi permettant d'engager avec vous une discussion approfondie sur chacune de ces mesures. Au-delà du seul bilan de leur mise en oeuvre, l'examen de ce texte aurait été l'occasion de débattre, ensemble, des éventuelles adaptations de notre cadre juridique à l'évolution de la menace. Les services de renseignement y étaient prêts. Le ministère de l'intérieur, le ministère des armées et l'ensemble du Gouvernement y étaient prêts. la mobilisation nationale rendue nécessaire par la gestion de la crise sanitaire y a fait obstacle. Le contexte n'a pas permis aux débats, dans chacune des chambres du Parlement, de se tenir de manière sereine. À ce contexte épidémique est venu s'ajouter l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 6 octobre dernier, sur le régime de conservation des données par les opérateurs de télécommunications. Les juridictions nationales tireront toutes les conséquences de cette décision européenne. Il nous faudra pouvoir en éclairer le Parlement et examiner avec lui les conséquences potentielles qu'il conviendrait d'en tirer dans la loi. Les sujets dont nous parlons sont majeurs pour la sécurité des Français. Ils touchent aux libertés fondamentales. Ils méritent d'être discutés avec tous les éclairages nécessaires. Aussi, compte tenu de la sensibilité et de la complexité des dispositions en question, il a semblé opportun au Gouvernement de proroger de quelques mois ces dispositifs pour réserver la tenue d'un débat de fond serein. En tout état de cause, la prolongation de l'expérimentation ne nous empêche pas- n'empêche pas nos services -de travailler. La mobilisation du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme est très forte. Elle se traduit, avec le soutien du Parlement, par une augmentation des moyens mis à la disposition des services spécialisés en matière de lutte antiterroriste, notamment les services de renseignement. Au total, 1 000 postes supplémentaires ont été créés depuis l'élection du Président de la République.

La lutte contre le terrorisme exige en effet de nous une mobilisation totale. Sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, avec l'engagement de l'ensemble des forces de sécurité et des services de renseignement, avec l'appui de la justice, M. le ministre

C'est pour ces considérations d'efficacité, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que je vous présente aujourd'hui, au nom du Gouvernement, ce projet de loi de prorogation. La parole

en matière de lutte contre le terrorisme, la convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat est habituellement de mise ; il est rare que députés et sénateurs ne parviennent pas à un accord pour doter les services de sécurité des moyens et des outils adéquats pour combattre ce fléau qui continue de frapper tragiquement notre pays de manière régulière. C'est pourquoi je regrette beaucoup que la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 22 octobre dernier pour examiner le projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen ne soit pas parvenue à un accord.

qu'il s'agisse des mesures issues de la loi SILT ou de la disposition de la loi relative au renseignement portant sur la technique de l'algorithme. En revanche, comme vous l'avez relevé, madame la ministre, nous avons une divergence profonde de méthode et de calendrier. Depuis le début de la navette parlementaire, le Gouvernement et les députés se cantonnent à l'idée de procéder à une prorogation « sèche », c'est-à-dire sans modification, des mesures de la loi SILT, ainsi que de la technique de l'algorithme. En première lecture, le Sénat a validé cette position pour la technique de l'algorithme, le temps qu'une réforme plus large de la loi relative au renseignement puisse être soumise à notre examen. En revanche, nous avons jugé que la prorogation sèche des dispositions de la loi SILT était non seulement injustifiée, mais également tout à fait inopportune au regard du niveau de la menace terroriste sur notre territoire. C'est pourquoi nous avons considéré comme essentiel, non seulement de pérenniser immédiatement ces mesures, mais aussi de leur apporter plusieurs ajustements afin de les rendre pleinement efficaces. Il s'agissait, premièrement, d'étendre le champ de la mesure de fermeture administrative aux lieux connexes aux lieux de culte, afin d'éviter le déport des discours radicaux vers d'autres lieux bien repérés par nos services secrets deuxièmement, de renforcer l'information des autorités judiciaires sur les Micas, de manière à assurer une parfaite articulation avec les mesures judiciaires telles que le contrôle judiciaire enfin, troisièmement, d'élargir les possibilités de saisie informatique dans le cadre d'une visite domiciliaire, dans les cas où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux données présentes sur un support ou un terminal informatiques.

la garde, mais faire preuve de réactivité pour doter nos services de sécurité des outils nécessaires pour assurer réellement la sécurité des Français. C'est la position que nous avons tenue en et que les députés ont catégoriquement refusé de suivre. À quoi sert donc d'expérimenter si l'on ne peut pas, à l'issue de l'expérimentation, pérenniser ? Nous regrettons que l'Assemblée nationale n'ait pas fondamentalement dévié de sa ligne en nouvelle lecture, alors même que l'actualité aurait dû l'amener à infléchir sa position. Sur la question de l'algorithme, il est heureux qu'elle se soit ralliée au Sénat, en acceptant de porter la nouvelle échéance de la technique au 31 décembre 2021, plutôt qu'au 31 juillet. C'est une bonne chose, car, avant de réformer la loi Renseignement, il nous faut laisser aux administrations de l'État le temps de tirer les conséquences des récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, qui risquent de remettre en cause le fonctionnement de plusieurs techniques de renseignement.

pourtant rappeler que les dispositions dont nous parlons font l'objet d'une évaluation régulière ? Le président de la commission des lois et moi-même, en tant que rapporteur, avons reçu toutes les semaines l'ensemble des arrêtés relatifs à ces dispositions sur notre territoire. Nous avons

Vous indiquez par ailleurs, madame la ministre, que votre texte n'affaiblit pas la lutte contre le terrorisme, car les mesures seront maintenues dans l'attente de leur pérennisation. Mais, ce faisant, vous écartez toute possibilité de leur apporter les ajustements que les services de votre ministère eux-mêmes estiment pourtant indispensables pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Vous ne pouvez pas en même temps déclarer vouloir faire une guerre sans merci aux djihadistes aux djihadistes et refuser de pérenniser définitivement dans la loi des mesures qui ont fait leurs preuves. Vous ne pouvez pas en même temps refuser notre proposition d'étendre la mesure de fermeture administrative aux lieux connexes aux lieux de culte dans lesquels agissent les prêcheurs de haine et défendre, comme s'y emploie le ministre de l'intérieur, une ligne ferme contre les discours séparatistes et lancer une offensive médiatique contre les mosquées où sévissent des discours haineux. Il y a là un manque profond de cohérence de la part du Gouvernement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission des lois a donc souhaité rétablir son texte de première lecture, afin de laisser une nouvelle possibilité au Gouvernement et à l'Assemblée nationale de se rallier à sa position,

de quatre mesures de sécurité publique centrées sur la lutte antiterroriste : les périmètres de sécurité, les fermetures de lieux de culte, les visites domiciliaires et les mesures individuelles de contrôle Nous constatons- je rejoins entièrement le propos du rapporteur Marc-Philippe Daubresse -que ces mesures ont été efficaces et qu'elles ont été mises été efficaces et qu'elles ont été mises en oeuvre sous un contrôle juridictionnel satisfaisant, qu'il s'agisse du juge administratif ou du juge judiciaire.

alors que la majorité sénatoriale souhaite qu'elles soient immédiatement pérennisées avec quelques ajustements- point sur lequel, je pense, il n'y a pas de désaccord. C'est donc évidemment dommageable,

-à ce que les États, pour des raisons de sécurité ou de justice, imposent aux opérateurs une obligation généralisée et indifférenciée de conservation des données. Il va donc falloir que, à l'intérieur de ce cadre jurisprudentiel, nous trouvions le moyen de faire fonctionner les algorithmes dont nos services ont besoin. Il est entendu que ce débat doit se conclure sur l'amélioration et l'extension du cadre légal du renseignement avant la fin de 2021. De toute manière, s'il doit y avoir, comme le préconise la commission, des améliorations en ce qui concerne par exemple l'étendue du pouvoir de fermeture de sites religieux, nous n'aurons pas longtemps à attendre pour constater un accord sur le fond.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 31 décembre 2020, un certain nombre de dispositions du code de la sécurité intérieure arriveront à échéance, si le législateur n'intervient pas. Dans ces conditions, nous comprenons bien évidemment la nécessité de sécuriser juridiquement des mesures qui pourraient intervenir au-delà de cette date, même si nous regrettons que le Parlement n'ait pas réussi à s'accorder sur les moyens d'y parvenir. Certes, si chacune des positions retenues se justifie, il est nécessaire de mener un débat approfondi sur les mesures de la loi SILT, son objet étant trop sensible pour être traité avec une quelconque forme de légèreté. C'est dans ce cadre que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer notre inquiétude et nos réserves s'agissant de la technique des algorithmes. Ce sujet doit être traité avec les précautions qui s'imposent, la seule poursuite d'une expérimentation en la matière peut faire l'objet d'un consensus. Cependant, nous pensons que les dispositifs expérimentaux, tout comme les dispositifs d'exception, ne doivent pas se multiplier au sein de notre législation. La période actuelle nous impose trop souvent d'y recourir, qu'il s'agisse de l'état d'urgence sanitaire et de ses mesures de police administrative ou bien encore du report du calendrier électoral. Certes, il y a des cas où l'urgence de la situation justifie qu'il faille procéder ainsi, mais il y en a d'autres pour lesquels nous donnons le sentiment de fuir nos responsabilités. Le Parlement écrit la loi, et l'essence de celle-ci n'est pas d'être qu'une mesure temporaire. Si, en 2017, il a été considéré comme nécessaire de sortir de l'état d'urgence, en même temps que de maintenir un certain niveau de sécurité, ce fut par l'application relais d'une nouvelle loi, non plus d'urgence, mais d'exception, dont les dispositions demeuraient, par leur contenu, limitées dans le temps. Nous voilà désormais à l'heure du bilan, et les circonstances nous imposeraient d'attendre encore. Il va sans dire que les objectifs du projet de loi dont nous discutons sont évidemment fondamentaux et essentiels, puisqu'il y est question des conditions d'exercice de nos libertés fondamentales. Nul ne souhaite discuter comme d'une formalité un texte ayant trait à la mise en place de périmètres de protection, à la fermeture de lieux de culte, à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ou à des visites domiciliaires et à des saisies. Nous entendons l'argument consistant à dire qu'il faut un débat et une réflexion, que la crise sanitaire n'a pas permis. Reste qu'il faut aussi entendre l'appel qui est fait, à savoir travailler à pérenniser les dispositifs, les ancrer durablement dans notre droit, voire les écarter s'ils ne convenaient pas, mais, du moins, qu'ils ne soient pas seulement « applicables jusqu'à une date » que l'on repousserait inlassablement. Un tel mode de fonctionnement ne serait pas satisfaisant. Il l'est d'autant moins que les bilans existent déjà. La mission pluraliste créée à cette fin par la commission des lois, en 2017, a conclu en faveur de la pérennisation des quatre dispositions temporaires, tout comme le Conseil constitutionnel, qui, à l'occasion de deux QPC, a jugé conforme à la Constitution l'essentiel des quatre mesures temporaires que nous évoquons. Nous ne pourrons pas proroger inlassablement les dispositifs, sauf à renoncer à ce que notre droit bénéficie d'une forme de stabilité. Mais vous comprendrez que la raison s'impose au groupe du RDSE, qui votera donc majoritairement en faveur de ce texte. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour comprendre ce dont nous débattons aujourd'hui en nouvelle lecture, il me semble nécessaire de revenir un instant sur l'origine des principales dispositions que comporte ce projet de loi, sans faire d'erreur sur les dates.

que la prorogation pure et simple reste la solution la moins pire, ou du moins la plus démocratique, en ce qu'elle permettrait un débat de fond sur ces mesures plus que problématiques à notre sens. En effet, de quoi s'agit-il ? Il est demandé à la représentation nationale de proroger, en procédure accélérée- sans bilans détaillés et exhaustifs de l'efficacité de nos outils législatifs de lutte contre le terrorisme des mesures préventives ordonnées sur la base de simples soupçons, restrictives de libertés, décidées par l'autorité administrative et soustraites, pour la plupart, au contrôle judiciaire. judiciaire. Si la loi SILT a transformé les assignations à résidence en mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les perquisitions en visites et saisies, il s'agit bien- ne nous y trompons pas -des mêmes mesures liberticides que celles de l'état d'urgence, qui contournent la justice pénale ordinaire et les protections qui lui sont associées. Je ne reviendrai pas sur les différents arguments que nous avons développés en première lecture pour vous démontrer l'inefficacité, en plus de leur dangerosité, de ces mesures. Mais je continue de m'étonner de la logique qui prévaut dans cette inflation législative, qui a pourtant fait les preuves de son échec. nous venons encore d'essuyer cette année plusieurs attentats terroristes, dont celui qui a été commis à l'encontre de Samuel Paty, le plus terrifiant sans doute, car dirigé contre tout notre modèle éducatif et la liberté d'enseigner ; celui perpétré à la basilique de Notre-Dame de Nice n'en est pas moins atroce. Mes chers collègues, nous pouvons être d'accord sur un point

Ces trente dernières années, seize lois ont été adoptées contre le terrorisme, auxquelles s'ajoutent trente-deux lois de lutte contre la délinquance, la plupart s'attaquant davantage à réduire nos libertés, sous couvert de sûreté, qu'à enrayer véritablement le terrorisme. Ainsi, le problème perdure Ne s'agirait-il pas à présent de faire le point sur notre stratégie en matière de lutte contre le terrorisme ? Il faudrait repenser, avec la hauteur de vue qui devrait être la nôtre, ce qui nourrit le terrorisme comme les relations commerciales et diplomatiques que Paris entretient avec certains pays complaisants à l'égard de ceux qui nous portent atteinte. Pour ce qui est de notre territoire national, les services de renseignement doivent être renforcés humainement et pas uniquement sur la base d'outils algorithmiques insensés ou pas. Notre police doit retourner au contact de nos concitoyens, non seulement pour y faire de la prévention, mais aussi pour remonter les informations nécessaires aux services de renseignement. Quoi qu'il en soit, un débat digne de ce nom doit se tenir sur le sujet, et l'échec des mesures dont il est question aujourd'hui doit être rapidement constaté, pour passer à la suite.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

là quelques surprises ... S'agissant des ajustements qui avaient été proposés par le Sénat sur l'information des autorités judiciaires, je ne suis pas sûr que cela change grand-chose. En revanche, l'extension du champ des mesures de fermeture administrative

semble manquer, à ce jour, une analyse comparative entre les besoins de nos services de sécurité et les conséquences à tirer de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un arrêt dont on ne mesure pas totalement les conséquences., il ne laisse pas de marges,

Cependant, dans la sauvegarde de la sécurité nationale, doit-on y intégrer les éléments de lutte contre le terrorisme ? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Il me semble donc que cet arrêt

de l'accord sur l'article 2 du projet de loi initial, nous n'aurons plus à nous prononcer sur la question des algorithmes. Permettez-moi cependant, en prévision d'une loi plus importante sur le renseignement qui nous est annoncée pour l'année prochaine, de formuler quelques remarques, car il s'agit à la fois de contraintes et d'enjeux européens et de la crédibilité de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Premièrement, la loi sur le renseignement prévoyait, du code de la sécurité intérieure, qu'un décret en Conseil d'État soit pris pour définir les conditions d'échange entre les différents services de sécurité et les administrations de toutes les informations en matière de données de connexion qui pourraient être récupérées. Or ce décret n'a jamais été pris,

spécifiquement dédié à délivrer des autorisations à la DGFiP. Cela pose un problème : d'un côté, on crée une CNCTR qui doit centraliser les demandes

soient mises en oeuvre dans des conditions respectant les libertés et l'intimité de chacun. La CNCTR doit donc être au coeur de nos préoccupations si nous souhaitons pouvoir garantir les libertés. garantir les libertés. Or un certain nombre de choses ne sont aujourd'hui pas parfaites de ce point de vue et mériteront d'être évoquées lors de la prochaine loi sur le renseignement- nous avions déjà déposé certains amendements sur le sujet. Enfin, il y a la

poserait problème. Il faut donc probablement réfléchir à une évolution du droit européen, car nous pouvons regarder comment les choses peuvent se faire à droit européen constant, même s'il n'est pas évident que cela soit possible.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme beaucoup de pays en Europe, la France fait face depuis de nombreuses années à une menace terroriste d'une particulière gravité. Nos forces de sécurité sont à pied d'oeuvre pour empêcher la réalisation de cette menace, nous saluons leur engagement. Malheureusement, et malgré leur travail, le risque ne peut jamais être totalement éliminé. Dernièrement, la France a ainsi été frappée à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. Nous saluons la mémoire des victimes. La vague de haine qui a traversé certains pays à l'occasion de la publication des caricatures laisse penser que cette menace terroriste ne va pas diminuer avec le temps, bien au contraire. Pour assurer la sécurité des Français, nous devons nous attaquer aux multiples racines de la mouvance terroriste. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République sera l'occasion d'apporter une réponse aux aspects idéologiques de la menace. Le texte que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture participe ainsi à la lutte contre le terrorisme. Il consiste en effet à proroger plusieurs dispositions, intéressant notamment nos services de renseignement. Si elles sont jugées utiles par ceux qui en font usage, ces mesures suscitent néanmoins des inquiétudes s'agissant des risques qu'elles sont susceptibles de faire peser sur les libertés individuelles et publiques. Ces dispositions ont donc été assorties d'un caractère temporaire, afin que leur maintien dans le droit commun soit réexaminé. Le délai fixé à cette occasion expire à la fin du mois. Nous regrettons que la commission mixte paritaire n'ait pas pu aboutir, dans la mesure où les positions défendues par chacune des deux assemblées du Parlement sont proches. Un consensus sur l'utilité des mesures en cause semble en effet se dessiner. La commission des lois a ainsi pu rappeler que, malgré l'échec de la commission mixte paritaire, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas de divergence sur le fond. La question qui demeure est celle de savoir s'il convient d'envisager une simple prorogation de ces dispositions ou bien s'il convient de les entériner sans attendre. La crise sanitaire a bouleversé le calendrier parlementaire : le projet de loi sur les mesures de lutte contre le terrorisme n'a pas pu être présenté au Parlement l'été dernier. Si la crise la crise sanitaire bouleverse le calendrier parlementaire, elle ne freine cependant pas la menace terroriste, comme l'a tristement rappelé l'actualité récente. C'est en ce sens qu'il nous apparaît important de soutenir la position défendue par notre rapporteur. Le groupe Les Indépendants considère en effet que l'urgence de la menace nous commande d'intégrer les ajustements proposés par le texte de la commission. Nous attendons avec impatience de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, un texte plus complet sur les mesures de lutte contre le terrorisme. Ces sujets sont cruciaux pour la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour leurs libertés.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'objectif de ce texte est, dans la continuité de la loi SILT de 2017, de proroger dans le droit commun des mesures d'exception, actuellement appliquées à titre expérimental. Ces dispositions, attentatoires aux libertés individuelles, ainsi qu'au respect de la vie privée, revêtaient pour l'heure un caractère temporaire. En 2017, le législateur avait ainsi estimé raisonnable de limiter leur application au 31 décembre 2020. L'échéance arrivant à son terme, l'exécutif s'est tout naturellement saisi de cette question. Deux choix s'offraient à lui : l'abrogation, si la représentation nationale estimait que ces dispositifs n'avaient pas fait leurs preuves leur pérennisation si, au contraire, l'efficacité de telles mesures pour la sûreté de nos concitoyens avait été démontrée. À ces options légitimes, le Gouvernement a préféré une troisième voie, la prorogation de ces dispositifs, estimant que la crise sanitaire pourrait être de nature à biaiser les discussions parlementaires.

Ainsi est-il proposé à l'article 1 de proroger de sept mois les dispositions de la loi SILT conférant à la police administrative selon nous trop importants, notamment ceux de déclarer la fermeture temporaire des lieux de culte, d'ordonner des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, ainsi que de réaliser des visites domiciliaires. Dans son article 2, le projet de loi prévoit une prorogation similaire de l'expérimentation des algorithmes votée en 2015 et prolongée en 2017. Ceux-ci permettent notamment de détecter les menaces terroristes les réseaux internet et de téléphonie mobile. En première comme en nouvelle lecture, le Sénat a souhaité non pas proroger, mais pérenniser les mesures prévues à l'article 1. Cette décision n'a semble-t-il pas fait l'unanimité en commission mixte paritaire, puisque celle-ci n'a pas été conclusive. Pour le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires, ni la pérennisation, par ailleurs rétablie en commission des lois par M. le rapporteur, ni la prorogation ne sont des solutions dans la mesure où nous nous opposons à l'intégration dans le droit commun de ces mesures de police administrative, qui ne sont pas anodines. Comment accepter que la loi française bascule dans une dimension si sécuritaire, faisant la part belle au soupçon, à l'arbitraire, aux dérives, à la stigmatisation par l'administration, au détriment de tout contrôle du juge judiciaire ? Comment accepter le recours aux algorithmes, alors que, entre 2017 et 2018, ceux-ci n'ont permis d'identifier que dix personnes à risque et alors qu'aucune d'elles ne présentait un danger sérieux pour la sécurité nationale ? En l'attente de dispositifs algorithmiques plus sophistiqués, susceptibles de nous apporter des résultats plus probants, il est préférable que nous privilégiions la dotation massive de nos services de renseignement en moyens humains et financiers. réel débat démocratique ni de bilans sérieux, elles ne sauraient être ni prorogées ni pérennisées. Pour ces raisons, le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires votera, comme en première lecture, contre ce texte.

En effet, la mission de contrôle et de suivi de mise en oeuvre de la loi SILT créée ici au Sénat a révélé tant la pertinence que l'efficacité des dispositions issues de cette loi dès le mois de février dernier. Or les députés ont fait le choix de se limiter à une prorogation sèche de ces mesures. Les derniers attentats perpétrés sur notre sol montrent pourtant que l'urgence demeure vive en la matière. De nos lieux de culte à nos écoles, il n'existe plus de sanctuaire à l'abri de la menace islamiste. Selon les dernières données du ministère de l'intérieur, 294 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été prises jusqu'au mois de juin dernier, dont 63 sont aujourd'hui en vigueur. Par ailleurs, 167 visites ont été réalisées depuis le 1 novembre 2017. Ces chiffres témoignent du niveau encore élevé de la menace. De plus, quelque 60 % des Français partis faire le djihad entre 1986 et 2011 en Afghanistan, en Bosnie ou en Irak ont récidivé à leur tour, selon une récente étude du Centre d'analyse du terrorisme. Mes chers collègues, un islamiste engagé dans une action violente a toutes les chances de récidiver, nous le savons tous maintenant. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le Gouvernement est en train de perdre une occasion d'aller plus loin et d'agir plus fortement dans la lutte contre le terrorisme islamiste alors même que nous n'avons pas de divergences de fond. Concernant la prorogation des dispositions de l'article 1 à l'article 4 de la loi SILT, en lieu et place de la pérennisation que notre rapporteur propose depuis le départ, nous disons aujourd'hui encore que, face à un phénomène jusqu'alors inconnu, nous devons utiliser les armes qui ont démontré toute leur pertinence.

Le report est justifié par plusieurs décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne relatives au régime de conservation des données par les opérateurs. L'exécutif a fait savoir que les conséquences de ces décisions n'auraient pas encore été tirées dans le droit national. Ce report ne doit pas retarder notre lutte en matière antiterroriste. Ne manquons pas l'occasion de donner à ceux qui nous protègent des moyens d'action efficaces. Nous le devons à nos services de renseignement, à nos forces de sécurité intérieure et à l'ensemble des Français. Pour conclure, je tiens, au nom de tout notre groupe, à remercier notre rapporteur, Marc-Philippe Daubresse, pour l'excellente qualité de son travail. Pour toutes les raisons évoquées, et en dépit du fait qu'il aurait mieux valu pérenniser dans la loi les mesures plutôt que de les prolonger temporairement, les sénateurs du groupe Les Républicains voteront ce projet de loi, tel qu'il a été amendé par la commission des lois en nouvelle lecture. La discussion

la définition des périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les visites domiciliaires. Ces mesures arrivant à échéance le 31 décembre 2020, un débat parlementaire aurait normalement dû se tenir afin d'évaluer leur pertinence et leur proportionnalité. Faisant fi des principes démocratiques et du devoir d'information du Parlement, le Gouvernement a décidé de proroger ces dispositions, sans véritable évaluation de fond en la matière. La droite sénatoriale est allée encore plus loin, puisqu'elle a décidé, en commission, en première comme en nouvelle lecture, de pérenniser ces mesures en les incorporant définitivement dans le droit commun. Mes chers collègues, nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle décision. Les dispositifs introduits par la loi SILT donnent à l'administration des pouvoirs exorbitants, qui bafouent les droits de la défense et contournent le contrôle du juge judiciaire. La sécurité de nos concitoyens est primordiale, mais la lutte contre le terrorisme ne saurait être assurée par le biais de procédures administratives attentatoires aux libertés

du Gouvernement ? Madame la sénatrice Esther Benbassa, vous proposez de supprimer des mesures qui sont, à notre sens, essentielles pour lutter contre le terrorisme. Le législateur a veillé ménager un réel équilibre entre la nécessaire préservation de la sécurité publique face à la menace terroriste et les libertés fondamentales, que vous avez rappelées. Le Parlement y a d'ailleurs scrupuleusement veillé. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé et l'utilisation qu'en a fait le Gouvernement l'a démontré. Les autorités de police administrative font un usage de ces mesures qui est adapté et, nous semble-t-il, proportionné à la menace à laquelle nous sommes confrontés. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Je

Finalement, monsieur le rapporteur, il serait assez malicieux que cet amendement soit adopté et que le texte retourne à l'Assemblée nationale modifié par notre groupe,

introduites pour une durée limitée en 2017 et, d'autre part, qu'il puisse modifier ou compléter les dispositions en cause pour mieux les adapter à certaines situations ou combler certaines lacunes

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la répartition des sièges de conseiller à l'assemblée de Guyane entre les sections électorales

Derrière l'adaptation du droit électoral à la démographie guyanaise se pose aussi la question de l'accompagnement de ces dynamiques en termes d'infrastructures, de réseaux ou de carénage des services publics.

Monsieur le président, monsieur le ministre, Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est, vous le savez, un texte d'ajustement. Il l'est tout d'abord par son objectif : adapter le mode de scrutin de l'assemblée de Guyane à la réalité démographique que connaît le pays. par sa portée, limitée : le texte que nous examinons se contente pour l'essentiel de formaliser et de pérenniser les règles ayant présidé à la répartition actuelle des sièges entre sections.

Cette évolution du nombre des habitants sur le territoire se double d'une modification de leur répartition. En effet, l'augmentation démographique n'est pas uniforme ; elle est différenciée selon les territoires, donc selon les sections électorales. La dynamique démographique est ainsi concentrée sur l'ouest guyanais, sur Saint-Laurent-du-Maroni et, dans une moindre mesure, sur l'agglomération de Cayenne. Il est du rôle du législateur de tirer les conséquences de cette double évolution démographique. Lorsqu'il a déterminé le mode de scrutin pour les sièges de conseiller à l'assemblée de Guyane, le législateur a en effet prévu une clause de réévaluation de leur nombre lorsque la population guyanaise atteignait deux paliers, fixés à 250 000 et 300 000 habitants. Alors que le premier de ces deux paliers a été franchi et que le second devrait l'être très prochainement, la proposition de loi entend prévoir une solution pérenne et souple pour la répartition des sièges de conseiller à l'assemblée de Guyane. En l'état actuel du droit, la répartition des sièges entre sections est déterminée directement par la loi, qui prévoit une attribution minimale de trois sièges par section. Le mode de scrutin prévoit également une prime majoritaire de onze sièges à la liste arrivée en tête des suffrages, elle-même répartie entre les différentes sections par le législateur, qui a prévu l'octroi d'au moins un siège par section. La présente proposition de loi n'a pas pour objet une nouvelle répartition temporaire des sièges, vouée à l'obsolescence après quelques années en raison des évolutions démographiques rapides que connaît la Guyane ; elle vise à instituer un mode pérenne de répartition des sièges. Il s'agit donc non pas de modifier le nombre de sièges par section, mais d'inscrire de manière pérenne dans la loi les règles de répartition des sièges entre les sections, de celles-ci à un arrêté du préfet de Guyane avant chaque scrutin. Dans le détail, la répartition s'effectuerait proportionnellement à la population de chaque section selon la règle de la plus forte moyenne. Chaque section se verrait attribuer, comme aujourd'hui, au moins trois sièges, afin d'assurer la représentation équitable et pluraliste des territoires. La prime majoritaire actuelle serait maintenue et répartie proportionnellement à la population de chaque section, selon la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d'un siège par section, conformément à la pratique actuelle.

que de la formalisation et de la pérennisation de la répartition actuelle, tout en renvoyant à un acte réglementaire la mise en oeuvre effective de ces règles. La proposition de loi, qui s'inscrit dans la continuité du dispositif existant et introduit une souplesse procédurale bienvenue, ne semble poser aucune difficulté de fond. Mes travaux ont donc consisté à m'assurer, d'une part, de l'accord politique sur le texte de l'ensemble des élus concernés et, d'autre part, de sa solidité juridique. J'ai ainsi consulté autant que faire se peut dans le calendrier contraint qui m'était imposé les élus concernés par la présente proposition de loi. Après avoir entendu Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane, Lénaïck Adam, député de Guyane et auteur de la proposition de loi, ainsi que mes collègues Georges Patient et Marie-Laure Phinera-Horth, j'ai acquis la certitude que le travail de concertation mené sur cette proposition de loi avait permis de faire émerger un consensus sur sa rédaction. Cela n'exclut aucunement les débats dont peut faire l'objet le mode de scrutin retenu par le législateur. Je pense en particulier à la question de la prime majoritaire, qui a été évoquée en commission. en commission. Néanmoins, pour légitimes qu'ils soient, de tels débats excèdent par leur portée le champ de la présente proposition de loi. Je note surtout qu'aucun des élus de terrain auditionnés lors de mes travaux préparatoires n'a évoqué de difficulté de fond sur le dispositif de la proposition de loi, préférant au contraire- j'y reviendrai -mettre l'accent sur la nécessité de son adoption rapide pour garantir la bonne tenue des élections. Mes travaux m'ont aussi permis de m'assurer de la solidité juridique du texte. Constatant que certaines harmonisations rédactionnelles devaient lui être apportées, j'ai ainsi proposé à mon homologue à l'Assemblée nationale, Lénaïck Adam, certains amendements, dont l'adoption par les députés a permis d'apporter des clarifications bienvenues dans la rédaction de la proposition de loi.

Ceux-ci se sont néanmoins inscrits dans un contexte particulièrement contraint. Comme vous le savez certainement, conformément au rapport de Jean-Louis Debré relatif à l'organisation des élections départementales et régionales, les élections pour l'assemblée de Guyane pourraient être maintenues au mois de mars 2021 si des différences objectives dans la situation épidémiologique le justifiaient. Dans ces conditions, et alors que le dispositif de la proposition de loi prévoit que le préfet de Guyane arrête la répartition des sièges avant le 15 janvier, le Parlement se voit contraint d'adopter la proposition de loi avant le 31 décembre. Cela implique, comme vous le savez, l'adoption du texte par un vote conforme du Sénat. Bien que je regrette ce calendrier contraint, j'en ai pris acte et j'ai engagé mes travaux en amont de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. En collaboration étroite avec M. Adam, nous avons mené un travail de fond permettant d'identifier et de corriger dès son examen à l'Assemblée nationale les quelques difficultés rédactionnelles que posait le texte, créant les conditions d'une adoption sans modification de la proposition de loi. Tel qu'issu des délibérations de l'Assemblée nationale, le texte me semble donc équilibré politiquement et solide juridiquement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au mois de mars prochain, les Guyanaises et les Guyanais devront se rendre aux urnes aux fins de renouveler leur assemblée. Mais, comme cela a déjà été indiqué dans les propos liminaires de notre rapporteure, dont je salue le travail, il nous faut réviser au préalable différentes dispositions dispositions en vigueur dans notre code électoral pour le bon déroulement de ce scrutin, et ce pour plusieurs raisons., parce que les circonstances l'imposent. En effet, l'accroissement de la démographie locale rend inapplicable la conciliation des articles L. 558-2 et L. 558-3 du code électoral. Si le nombre de conseillers augmente mécaniquement, il nous appartient de revoir leur répartition au sein des différentes sections électorales de la circonscription. Au demeurant, nous voulons nous féliciter du consensus qui a pu s'exprimer dans la préparation de ce texte, tant au Parlement qu'avec les autorités guyanaises et les élus locaux. Si les ajustements des conditions de scrutin sont parfois observés d'un regard suspicieux, par crainte qu'ils consistent en une manoeuvre pour orienter le résultat final, ce texte est au contraire salué comme une avancée., une avancée., car la rédaction actuelle ne permet que dans une faible mesure de s'adapter au changement de circonstances de fait, comme, par exemple, le dynamisme démographique que connaît justement la population de Guyane. En l'état actuel du droit, il est nécessaire de légiférer à chaque évolution. Or, comme l'a indiqué l'Insee en 2019, le nombre d'habitants sur le territoire guyanais a dépassé les 280 000, de sorte qu'en dix ans la population s'est accrue de près de 30 %. Ainsi, la grande vitalité démographique du territoire guyanais, si elle persiste, nous obligerait à légiférer de nouveau très rapidement. Aussi, il apparaît judicieux de repenser le système actuel, afin de limiter autant que faire se peut tout foisonnement législatif excessif. Je salue ainsi le dispositif proposé, qui consiste en une répartition des sièges entre les sections proportionnellement à leur population. C'est un mode de calcul qui n'appelle pas de contestation. De ce point de vue, il apparaît plus sensé que cette répartition soit arrêtée par le représentant de l'État en Guyane, suivant un mode de calcul fixé par la loi, plutôt qu'elle soit directement inscrite dans la loi avec l'inconvénient majeur de devoir légiférer de nouveau, comme je l'indiquais précédemment.

La proposition dispose que la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, quand les onze sièges du droit en vigueur représentaient environ 21 % du nombre total de sièges. Le nouveau dispositif sera donc insensible du point de vue des institutions, tout en permettant une simplification du droit et un allégement de la production législative à venir. Il y a donc lieu de s'en féliciter. Au-delà des seules considérations de mécanique juridique, nous devons garder à l'esprit que les changements démographiques en Guyane vont avoir des conséquences puissantes dans les années à venir. S'il y a bien sûr la question du poids de l'immigration illégale, il faut dire un mot, à quelques jours de l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 et de la présentation de la loi confortant les principes républicains, de certaines difficultés auxquelles la démocratie locale guyanaise est confrontée, avec une montée en puissance de dérives religieuses et communautaristes. Si la Guyane connaît un régime spécifique en matière de laïcité, cette singularité ne doit pas nous conduire à demeurer passifs, quelles que soient les dérogations qui ont pu être accordées au fil de l'histoire. À cette occasion, je voudrais saluer l'initiative du groupe CRCE, qui a déposé une proposition de loi en ce sens le 6 novembre dernier ; je me permets d'encourager nos collègues à l'inscrire prochainement à l'ordre du jour de nos travaux.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la présente proposition de loi fait consensus : c'est un sujet technique et pratique, circonscrit à l'assemblée de Guyane, mais permettant d'assurer le bon fonctionnement de cette institution démocratique. Ce texte relève d'un impératif démocratique urgent, car ses dispositions ont vocation à s'appliquer aux prochaines élections, prévues pour le mois a été particulièrement bousculé en Guyane, ces élections pourraient y être maintenues, et le rapport de Jean-Louis Debré conseille de réaliser une évaluation spécifique pour cette collectivité. Plus que d'adapter le nombre de conseillers au regard de l'évolution démographique en Guyane, ce texte propose d'inscrire dans la loi les règles de calcul pour définir leur nombre et les répartir, afin de ne pas avoir à passer par une nouvelle loi, alors que le second seuil de 299 999 habitants pourrait être rapidement dépassé, amenant le nombre de conseillers à soixante et un. Le représentant de l'État établira cette répartition avant chaque échéance électorale en suivant les règles fixées dans la loi, pour le nombre de conseillers de chacune des huit sections comme pour la prime majoritaire. Si la vitalité démographique de la Guyane nous amène à faire évoluer la représentation de cette collectivité, nous regrettons qu'elle ne soit pas également à l'origine de l'augmentation des moyens fléchés En dix ans, la population y a augmenté de 10 %, avec un taux de natalité de 26,4 ‰, soit plus du double des autres départements français. Cela a des conséquences sur le quotidien des Guyanais en termes d'infrastructures, de services publics et plus globalement de qualité de vie.

La situation sanitaire en Guyane est alarmante. L'épidémie a révélé les défaillances structurelles du système de santé, aggravées par la pauvreté et la précarité de la population. Alors que 45 % de la population guyanaise vit dans un désert médical, le manque d'anticipation a été de mise face à la non-prise en compte de ces réalités, et la population en paye le prix. Pourtant, en 2017, les mouvements de protestation guyanais alertaient sur l'état déplorable des hôpitaux, le manque de personnel ou encore la encore la vétusté des réseaux d'approvisionnement d'eau. L'étude réalisée cet été par des associations, le centre hospitalier et l'ARS de Guyane chiffre le niveau d'insécurité alimentaire qui existe dans certains quartiers : deux ménages sur cinq ont eu une alimentation insuffisante sur une semaine, plus de 80 % ont souffert de la faim dans le mois et la crise a dégradé le budget des ménages, qui, pour la moitié, disposent de 30 euros ou moins sur une semaine pour nourrir l'ensemble d'un ménage. Pour reprendre les mots de Solène Wiedner-Papin, directrice de la santé publique de l'ARS : « Les données sont effrayantes. L'évolution de la population joue également sur la jeunesse guyanaise, puisque les moins de 20 ans représentent 40 % de la population ; c'est le deuxième département le plus jeune de France, après Mayotte. Tout comme pour la santé, la collectivité figure au 123 rang mondial pour l'éducation, accusant un écart inacceptable avec la métropole. Les jeunes sont les premiers touchés par la pauvreté, renforcée par l'actuel ralentissement économique, dans une collectivité où une personne sur cinq est touchée par l'illettrisme et où les écoles sont saturées dès la maternelle. Chez les 25-29 ans, seuls 58 % des Guyanais sont en activité, contre 86 % en métropole. Le manque de diplômés et d'attractivité de la Guyane a aussi des effets sur la pénurie de personnels de santé. La Guyane n'a pas attendu la crise pour souffrir de tels maux. Des investissements considérables sont attendus, notamment dans le secteur public. Nous voterons cette proposition de loi, car c'est un texte de bon sens, mais nous souhaitions saisir cette occasion pour rappeler que les institutions démocratiques ont peu de consistance sans une égalité de droits et sans justice sociale pour les citoyennes et les citoyens.

en renvoyant à un arrêté du préfet de Guyane la mise en oeuvre de ces règles avant chaque scrutin. Cela nous paraît parfaitement adapté.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chacun le sait, le 24 janvier 2010, à plus de 57 %, les Guyanais ont approuvé par référendum la fusion du département et de la région que la création d'une collectivité unique régie par l'article 73 de notre Constitution. L'article L. 558-2 du code électoral

contre 11,1 ‰ dans l'ensemble des départements. La Guyane est aussi le territoire français le plus jeune, avec Mayotte, une personne sur deux étant âgée de moins de 25 ans.

Dans la mesure où le droit en vigueur prévoit une nouvelle répartition des sièges après le franchissement d'un autre seuil et vu le dynamisme démographique de la Guyane, une nouvelle modification législative serait nécessaire dans peu de temps.

La première portait sur le renvoi de l'application des règles d'attribution des sièges à un arrêté du préfet de Guyane, et non de M. le ministre de l'intérieur ou de M. le ministre des outre-mer. notre rapporteure, que je tiens à saluer, le renvoi au pouvoir réglementaire de la répartition effective des sièges ne présente pas de risque constitutionnel.

pour l'élection des assemblées locales constituent des composantes du régime électoral de celles-ci. En l'espèce, dans la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires le législateur a fixé le nombre de conseillers départementaux et encadré la compétence du pouvoir réglementaire pour la mise en oeuvre de ces règles. La rédaction retenue pour la proposition de loi prévoit donc la fixation de règles pérennes en matière de répartition des sièges entre les différentes sections électorales. Ce faisant, elle place le pouvoir réglementaire en situation de compétence liée et, par conséquent, il n'est pas utile de conférer au ministre de l'intérieur la charge d'adopter un tel acte.

En effet, il est important de souligner qu'un travail préalable a été effectué en commun avec l'Assemblée nationale sur ce texte. Depuis le 1 janvier 2016, la Guyane est une collectivité territoriale unique, qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région. Elle est dotée d'une assemblée unique chargée de régler, par ses délibérations, les affaires de la collectivité. Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans, au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Pour assurer une stabilité à cette assemblée, la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou arrivée en tête au second tour se voit attribuer une prime majoritaire de onze sièges. L'assemblée de Guyane est actuellement composée de cinquante et un conseillers, le nombre de sièges étant fixé selon la population de la collectivité

999 habitants. Or les estimations font état de plus de 290 000 habitants au 1 janvier 2020 : un premier seuil a donc été franchi et le second pourrait l'être prochainement, compte tenu de la vitalité démographique de ce territoire. Cette augmentation du nombre de conseillers, qui est automatique, n'est pas sans conséquence. En effet, la Guyane forme une circonscription unique, divisée en huit sections électorales. Le code électoral répartit les cinquante et un sièges de conseiller actuels par section. Cette répartition doit désormais être révisée pour tenir compte du passage à cinquante-cinq conseillers. Plutôt que d'effectuer un tel ajustement technique, il a paru pertinent d'aller plus loin, en inscrivant dans la loi la règle de calcul permettant la répartition des sièges. Un arrêté du représentant de l'État en Guyane en fera l'application. Cette règle est la suivante : les sièges sont répartis entre sections proportionnellement à leur population, en suivant la règle de la plus forte moyenne. En outre, chaque section dispose d'au moins trois sièges. Par souci de cohérence, cette évolution a été étendue à la prime majoritaire, car, en l'état du droit, aucune évolution de cette prime majoritaire n'accompagne l'augmentation du nombre de sièges de conseiller. remplacement du nombre onze, inscrit dans le code électoral, par une fraction constante, à savoir 20 % des sièges, apparaît comme une solution satisfaisante. Ainsi, le nombre de sièges octroyés au titre de la prime majoritaire passera automatiquement de onze à treize lorsque le nombre de conseillers atteindra à la suite du prochain franchissement de seuil de population. La répartition de ces onze, puis treize sièges entre les sections suivra la règle de calcul établie. Chaque section aura au moins un siège. Cette évolution présente un double intérêt. D'une part, nous n'aurons plus à intervenir à chaque franchissement de seuil démographique- l'adoption de deux lois successives pour un simple ajustement technique ne se justifie guère. D'autre part, le préfet pourra désormais actualiser la répartition par section à chaque renouvellement de l'assemblée, y compris lorsqu'aucun seuil de population n'aura été franchi, afin d'assurer une meilleure représentation de la population. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis du consensus qui s'est fait autour de cette proposition de loi, mais également de la prise en considération des réalités de la Guyane. Le groupe Les Indépendants votera à l'unanimité en faveur de ce texte. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi tend à valider l'augmentation du nombre de conseillers de l'assemblée de Guyane et à décider de la répartition des sièges Ce texte, déposé par Lénaïck Adam, député de Guyane, n'entraîne aucune modification du mode de scrutin des élections de la collectivité territoriale de Guyane, mais il permettra une meilleure représentation de la population au sein de cette collectivité. Il répond aux dispositions déjà prévues par le code électoral. Je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail fourni par les rapporteurs des deux chambres. Je remercie particulièrement notre collègue rapporteure, Catherine Belrhiti, qui a bien voulu nous auditionner. Elle a su saisir deux points qui me semblent essentiels : d'une part, le consensus de toute la classe politique guyanaise sur les objectifs visés par cette proposition de loi ; d'autre part, la nécessité d'une adoption rapide, pour une promulgation de la loi avant le 31 décembre 2020, condition indispensable pour que les élections de la collectivité territoriale de Guyane aient bien lieu au cours de l'année 2021, à l'instar des élections régionales et départementales. Ainsi, cette proposition de loi prévoit que la répartition du nombre de sièges par section, le nombre de sièges octroyés au titre de la prime majoritaire et la répartition par section de ces derniers devront être déterminés, en application des règles énoncées par la loi, par un arrêté préfectoral pris au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane. Mme la rapporteure et mes collègues ont su préciser les dispositions de cette proposition de loi, avec un excellent travail de coordination mené entre les deux assemblées. Je me permettrai donc, monsieur le ministre, de me faire le porte-voix de mes collègues guyanais sur un autre sujet, qui nécessite toute notre attention. Le texte qui nous réunit ici aujourd'hui trouve sa source dans l'évolution démographique de la population guyanaise. Comme vous le savez, en Guyane, la démographie est galopante. La Guyane est, après Mayotte, le département français dans lequel le taux de natalité est le plus élevé et le taux de mortalité le plus faible. À ces éléments, s'ajoute une pression migratoire constante et de plus en plus prégnante. La compilation de ces phénomènes nous pousse à interroger les chiffres du recensement effectué par les services de l'État. Comment expliquer aux Guyanais, qui voient pousser des bidonvilles et des squats sur les terrains vagues et dans les maisons abandonnées, que nous n'avons toujours pas franchi la barre des 300 000 habitants sur ce territoire aussi vaste que le Portugal ? Comment expliquer à mes compatriotes qu'avec nos 290 000 habitants nous produisons autant de déchets que 300 000 Nantais, alors que notre système de collecte est malheureusement défaillant, voire inexistant sur une large partie du territoire ? L'ancienne maire de la ville de Cayenne que je suis est plus que convaincue que les chiffres de la population en Guyane sont largement sous-estimés, et j'insiste sur ce terme.

En Guyane, l'organisation du recensement de la population s'appuie sur les mêmes textes réglementaires que pour le reste de la France. Les collectes sont exhaustives tous les cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants et annuelles, sur la base de 8 % des logements, pour les communes de plus de 10 000 habitants. Mais l'Insee et les communes doivent s'adapter davantage pour effectuer des collectes plus précises et en cohérence avec les particularités guyanaises. Je pense à la collecte dans l'habitat informel, dans les zones d'habitat où les naissances sont très rapides, comme en bord de fleuve et dans les zones d'orpaillage illégal. Malgré les efforts des uns et des autres, nous sommes encore loin du compte. Cette sous-estimation de la population a d'autres conséquences. Je rappelle ainsi que l'État se fonde sur ces chiffres pour calculer, notamment, la dotation globale de fonctionnement. Certes, la DGF est en progression en Guyane, mais elle demeure l'une des plus faibles de l'ensemble des collectivités ultramarines. Or elle est la première et principale source contributive au budget des communes de Guyane, compte tenu de la faiblesse des ressources fiscales. Les budgets des collectivités de Guyane peuvent donc se voir amputer de dotations, du fait d'une évidente sous-estimation de la population, qui sert de base au calcul de la DGF. Par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans cet hémicycle la situation des écoles de Guyane, qui ne peuvent pas scolariser l'ensemble des enfants se présentant à leurs portes, ce qui pose un véritable problème dans un territoire où nombre de jeunes se trouvent en déshérence.

que l'État et ses services déconcentrés assurent un recensement plus efficace et précis de la population de Guyane. Nous savons pouvoir compter sur les engagements du Gouvernement. Le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte, essentiel à la vie démocratique en Guyane. La discussion générale est